La séance est reprise. Mes chers collègues, en accord avec le Gouvernement et la commission, nous pourrions d'ores et déjà prévoir de lever notre séance de demain, vendredi 16 juillet 2021, à dix-sept heures. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. Par ailleurs, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mardi 20 juillet, après-midi et soir, de l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi dit « Climat et résilience », », sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, puis de la nouvelle lecture du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, et, enfin, de la suite de l'examen du projet de loi dit « 3DS Acte est donné de ces demandes. En outre, en raison de la tenue de la conférence des présidents à quatorze heures quinze, l'ouverture de la séance publique du mardi 20 juillet serait reportée à quinze heures. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. Le Gouvernement demande également que la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement soit inscrite à l'ordre du jour du mercredi 21 juillet, l'après-midi et le soir. Acte est donné de cette demande. Nous pourrions fixer le délai limite de dépôt des amendements de séance sur ce texte au mercredi 21 juillet, à l'ouverture de la discussion générale. De plus, afin de pouvoir terminer l'examen de ce texte mercredi, nous pourrions d'ores et déjà prévoir d'ouvrir la nuit du mercredi 21 juillet. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. Mes chers collègues, par la même lettre, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du jeudi 22 juillet, le soir, et du vendredi 23 juillet, le matin et l'après-midi, du projet de loi relatif à l'adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire. est donné de cette demande. Pour l'examen de ce texte, nous pourrions réserver la séance du soir du jeudi 22 juillet à la discussion générale. Nous pourrions également fixer le délai limite de dépôt des amendements de séance au jeudi 22 juillet, à l'ouverture de la discussion générale. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle le débat sur l'orientation des finances publiques et la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général du budget, madame la rapporteure générale de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, l'exécution budgétaire de l'année 2020 témoigne de la réponse massive et rapide que l'État a apportée pour soutenir les ménages, les entreprises et les collectivités locales face à une crise historique. Pour ce faire, et grâce à votre concours, nous avons donné à l'État les moyens d'être à la hauteur, par les différentes lois de finances rectificatives que le Gouvernement vous a proposées. de ces choix imposés par la crise, l'exercice 2020 a fait naître de nouveaux défis, auxquels nous ne pourrons répondre que par la croissance de l'économie et la poursuite des réformes. Il me semble utile de revenir tout d'abord devant vous sur l'ensemble des enseignements et défis que nous pouvons tirer de l'année 2020, puis d'évoquer la situation de 2021, et, enfin, de vous présenter les orientations que le Gouvernement propose pour les finances publiques de l'État pour l'année 2022.

À la suite de l'annonce du premier confinement, le Gouvernement a présenté au Parlement, dès le 18 mars 2020, un premier projet de loi de finances rectificative d'urgence, adopté cinq jours plus tard seulement. Ces délais d'examen resserrés ont apporté la preuve de l'esprit de concorde et de responsabilité que la crise a suscité et que nous nous sommes collectivement efforcés de maintenir depuis Cette première loi de finances rectificative, ou LFR, nous a permis de créer trois dispositifs de soutien, aujourd'hui bien connus de nos compatriotes. Ils ont depuis lors été adaptés et complétés par trois LFR successives et de nombreux autres textes législatifs et réglementaires. Grâce à votre vigilance et à l'attention des services de l'État, le soutien apporté a été enrichi, pour prendre en compte les spécificités sectorielles, réglementaires et géographiques de chacun des acteurs qui ont eu recours à ces dispositifs. Je pense, en premier lieu, à l'activité partielle. Forts de l'expérience des crises passées, notamment celle de 2008, nous avons mis en place un soutien massif pour protéger les entreprises, leurs salariés et leur savoir-faire, et, ainsi, préserver les compétences nécessaires à la reprise. Nous vous avons donc proposé une forme d'activité partielle très généreuse qui, depuis le début de la crise, a représenté un montant total d'environ 35 milliards d'euros, dont 26,3 milliards d'euros en 2020. Sur cette dernière somme, 17,8 milliards d'euros ont été décaissés depuis le budget de l'État, le reste étant pris en charge par l'Unédic. Au plus fort de la crise, en avril 2020, c'est 1 million d'entreprises qui a fait appel à l'activité partielle, pour plus de 8 millions de salariés. Je pense ensuite au fonds de solidarité. Si ce dispositif a d'abord été pensé comme un filet de sécurité à court terme pour les très petites entreprises, nous l'avons rapidement transformé en un soutien massif à destination de l'ensemble des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire. Depuis sa création, 31 milliards d'euros ont été versés en réponse à plus de 9,6 millions de demandes, dont 11,8 milliards d'euros et 6,3 millions de demandes pour la seule année 2020. Au total, quelque 2,2 millions d'entreprises ont pu bénéficier du fonds de solidarité. Les délais de versement des aides ont été, dans leur grande majorité, de trois jours ou moins. J'en profite pour remercier l'ensemble des administrations de Bercy, ont fait preuve d'une grande réactivité et d'un engagement sans faille pour mettre en oeuvre, conduire et adapter le fonds, qui a connu pas moins de onze versions en 2020, sans compter les dispositifs « cousins

les PGE n'ont pas maintenu en vie beaucoup d'entreprises « zombies ». Je puis vous dire que nous sommes particulièrement rassurés sur la capacité de remboursement des entreprises lorsque les échéances vont arriver. D'autres formes de soutien de l'État ont complété l'arsenal des aides, comme les reports fiscaux et sociaux, les exonérations de cotisations sociales, les aides au paiement ou encore le renforcement exceptionnel des participations financières de l'État au capital d'entreprises stratégiques. Le financement de ces dispositifs n'était pas un enjeu anodin. Nous avons toujours été prudents et nous avons toujours fait preuve de prévoyance, pour que jamais les crédits nécessaires Compte tenu de l'incertitude extrême dans laquelle nous a plongés la crise, nous vous avons proposé à plusieurs reprises d'ouvrir des crédits d'un montant suffisamment important pour faire face à d'éventuels durcissements de la situation sanitaire, ce qui s'est souvent justifié par la suite. Le Parlement et la Cour des comptes ont fait part de leurs interrogations légitimes quant au niveau des reports de crédits de 2020 vers 2021. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer devant vous lors de l'examen du PLFR 2021,

celle-ci a été limitée à 11 % en novembre 2020 et à entre 6 % et 7 % au mois de décembre 2020. Notre objectif était d'assurer le financement de l'urgence, tout en informant avec sincérité le Parlement.

verser, pour des questions de trésorerie, les aides aux entreprises qui les attendaient. Je crois que l'État a répondu de manière efficace et proportionnée à la crise. C'est le résultat que l'on peut afficher, plus d'un an après son déclenchement. Les dispositifs, qui ont évolué avec les connaissances sur la maladie et avec l'adaptation de notre société et de son économie, ont permis de préserver le pouvoir d'achat des Français. Celui-ci a globalement augmenté de 0,4 % en 2020, d'après l'Insee, et cela malgré la forte baisse de l'activité. de l'activité. Il faut souligner, notamment, que les revenus soumis à retenue à la source, c'est-à-dire essentiellement les salaires et les retraites, ont été supérieurs de 3,5 % en 2020 par rapport à 2019. Cette tendance se confirme au début de l'année 2021. Par ailleurs, les aides de l'État ont permis de préserver les entreprises, notamment les TPE et les PME, qui constituent la base de notre tissu économique, industriel et productif. Elles ont largement bénéficié de l'activité partielle et du fonds de solidarité, qui ont limité le nombre de faillites à un niveau historiquement bas, malgré la crise. Enfin, la capacité de financement des collectivités locales a été préservée. Elles affichaient le plus souvent une excellente santé financière à la fin de l'année 2020 : leur besoin de financement était de 1,2 milliard

Notre politique d'aide exceptionnelle face à la crise a donc montré son efficacité. Elle a permis à tous les acteurs économiques de reprendre leur activité de la manière la plus sereine et la plus dynamique possible. Je saisis l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour dire que, si nous avons pu mettre en place ce soutien efficace aussi promptement et massivement,

le ratio de dette publique a diminué en 2018, puis en 2019, pour les premières fois depuis 2007. Dans le même temps, nous avons tenu nos engagements en proposant au Parlement, qui a voté cette mesure, de baisser les impôts des Français, puisque le taux de prélèvements obligatoires a diminué de 1,3 point de PIB entre 2017 et 2019. C'est un élément sur lequel je souhaite insister, car j'ai la conviction que, sans le sérieux budgétaire dont nous avons fait preuve avant la crise, nous n'aurions pu réagir aussi fortement ni aussi efficacement. C'est aussi

qui a permis de maintenir les recettes fiscales à un niveau plus important que celui que nous envisagions. Elles sont supérieures, dans la loi de règlement que je vous propose d'adopter, de 6,7 milliards d'euros par rapport à la dernière prévision de la LFR 4

nous devons aussi nous pencher sur les orientations que nous vous proposons de retenir pour la préparation du budget 2022. Au-delà du seul budget de l'État, la sortie de la crise que nous espérons tous- de la crise épidémique, s'entend

si le déficit a été historique en 2020, à hauteur de 9,2 %, il restera très élevé en 2021, même si l'amélioration des perspectives de croissance nous permet de le revoir à la baisse,

Ce plan a des effets : la consommation est soutenue ; l'investissement des entreprises est fort. C'est ce qui nous permet de réviser notre hypothèse de croissance, initialement prévue à 5 %, jusqu'à 6 %, en lien avec les dernières estimations de l'Insee. Au-delà de cette relance rapide, le Président de la République a fait part de son intention de mettre en place un plan d'investissement pour construire la France de 2030, une France à la hauteur des défis d'aujourd'hui, renforcée par des industries à haute valeur ajoutée et au rendez-vous avec des innovations de rupture.

les modalités de financement, à une échelle nationale ou communautaire, mais aussi d'examiner ce qui relève de crédits budgétaires, de mobilisation d'outils comme le programme d'investissements d'avenir ou encore des dispositifs mis en place par la Banque publique d'investissement, Par ailleurs, le Président de la République s'est aussi prononcé pour la mise en place d'un revenu d'engagement, pour aider les jeunes sans emploi et sans formation à s'insérer dans le monde du travail, et ce grâce à un suivi personnalisé, dans une logique très équilibrée entre les droits et les devoirs. C'est un engagement sur lequel nous vous proposerons aussi de travailler d'ici à la présentation du projet de loi de finances pour 2022. En outre, ce projet de loi de finances pour 2022 doit être l'occasion de poursuivre nos efforts dans les domaines qui nous apparaissent prioritaires. Je pense à l'éducation, à la justice, à la sécurité, à l'environnement et au soutien aux plus fragiles. La crise ne nous a pas lié les mains, et le projet de loi de finances pour 2022 doit nous permettre de décliner d'abord les lois de programmation- je pense à la loi de programmation militaire, à la loi de programmation pour la justice

Nous poursuivrons aussi notre effort en matière de sécurité. Le ministère de l'intérieur verra ses moyens augmenter de plus d'un milliard d'euros, pour donner aux forces de l'ordre les moyens de mener à bien leur mission. Le ministère de la justice, pour la seconde année consécutive, verra les crédits dont il dispose augmenter de 8 %.

et que nous devons dégager des moyens pour accompagner la réforme et la modernisation de la justice. Nous maintiendrons aussi notre engagement pour l'éducation. Le Grenelle de l'éducation est d'ores et déjà décliné à hauteur de 700 millions d'euros, ce qui permettra de revaloriser les corps encadrants et enseignants, mais aussi de financer la protection sociale complémentaire pour la part relevant désormais obligatoirement de la participation de l'employeur. Nous poursuivrons le déploiement de l'école inclusive, avec le recrutement de 4 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap supplémentaires à la rentrée de septembre 2022.

et, conformément à l'engagement du Président de la République, le dispositif « 1 jeune, 1 solution » sera prolongé : il a déjà permis à 2 millions de jeunes de trouver une formation, de décrocher un emploi ou encore de signer un contrat d'apprentissage.

Toujours dans le projet de loi de finances pour 2022, que j'aurai l'occasion de présenter en conseil des ministres à la fin du mois de septembre prochain, nous continuerons d'investir massivement pour la transition écologique. Ainsi, l'enveloppe du dispositif MaPrimeRénov'sera abondée afin de relancer et d'accompagner la transition énergétique.

En somme, le virus n'aura pas fait vaciller nos ambitions, et nous ne dérogerons pas à nos engagements dans les années à venir. Autre engagement auquel nous sommes attachés : continuer à réformer, et cela en 2022. Nous continuerons en effet à transformer l'État et son action. La réforme de la fonction publique, par exemple, suivra son cours l'examen des derniers textes d'application. De plus, nous mettrons en oeuvre, évidemment, la réforme de la haute fonction publique annoncée par le Président de la République.

Ce sera le cas progressivement, comme nous l'avons dit, et nous prenons ainsi pleinement en compte l'importance de l'objectif de soutenabilité de nos finances publiques. En effet, si nous pouvons réviser l'hypothèse de croissance de 5 % à 6 %, il n'en reste pas moins que la trajectoire de nos finances publiques est dégradée

à un peu plus de cinq heures du matin, après que les derniers arbitrages ont été rendus. Les excuses que je présente à la représentation nationale pour cet envoi tardif se doublent de mes remerciements pour la mobilisation, nuit et jour, y compris les jours fériés, de mes équipes et de celles de la direction du budget.

de ne pas gâcher, d'une certaine manière, les efforts extrêmement importants que nous avons déployés pour faire face à la crise et accompagner la relance. En second lieu, nous allons continuer à travailler à la stabilisation des dépenses de fonctionnement. Cela se traduira notamment

Nous continuerons à mettre en oeuvre un certain nombre de réformes. Le Président de la République a rappelé sa volonté de mettre en place, dès le 1 octobre 2021, la réforme de l'assurance chômage. Par ailleurs, et peut-être de manière moins visible, nous travaillons à une refonte globale de la politique des achats de l'État,

Enfin, nous aurons l'occasion d'ouvrir plusieurs chantiers de réforme de la gouvernance des finances publiques, chantiers internes, notamment avec la réforme de l'organisation financière de l'État, la volonté de responsabiliser les gestionnaires publics, mais aussi le rapprochement des directions financières du ministère avec celles du contrôle budgétaire externe, qui est exercé par le ministère des comptes publics. chantier est partagé avec le Parlement, puisque c'est l'objet des propositions de loi organique déposées, d'une part, par Thomas Mesnier, et, d'autre part, par Éric Woerth et Laurent Saint-Martin, que l'Assemblée nationale aura à examiner la semaine prochaine. C'est aussi l'objet de la proposition de loi organique déposée par Mme la présidente Deroche et M. Jean-Marie Vanlerenberghe en matière de finances sociales. J'ai la conviction que cette réforme des lois organiques et du cadre dans lequel s'inscrit la gouvernance des finances publiques sera utile pour recouvrer de la lisibilité et rendre à notre niveau de dépenses

est de revenir à une forme de soutenabilité, donc à une normalisation des finances publiques et de leur gouvernance à l'échelle nationale. Nous voulons continuer à répondre à la crise et accompagner la relance, mais aussi financer les priorités du Gouvernement et du Président de la République, sans compromettre l'avenir.

et le respect de l'autorisation parlementaire, et à celui de l'avenir, avec le débat d'orientation de nos finances publiques pour 2022, qui s'accompagne d'un rapport préparatoire, dans lequel le Gouvernement présente la situation et les perspectives de l'économie pour les années à venir, en précisant sa stratégie en matière de finances publiques. Concernant, tout d'abord, l'exécution budgétaire de l'année 2020, on peut sans nul doute la qualifier « d'exceptionnelle », compte tenu bien sûr de l'épidémie de covid-19 et de ses conséquences sur l'économie mondiale.

Chacun le sait, cette crise a rendu urgente et vitale la mise en oeuvre de mesures de soutien, tant aux entreprises qu'aux ménages. Ainsi, les dépenses de l'État ont augmenté considérablement, avec en particulier plus de 40 milliards d'euros consacrés à la seule mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » qui n'existait même pas initialement.

à la fois d'une croissance supérieure à son potentiel et d'un fort dynamisme des prélèvements obligatoires. Mon prédécesseur Albéric de Montgolfier l'avait souligné dans cette même enceinte, et cela nous a fragilisés lorsque la crise est survenue. Fort heureusement, les conditions de financement sur les marchés financiers sont restées historiquement favorables. Ainsi, les administrations n'ont pas pu prendre à leur compte les pertes de revenus des entreprises dans des proportions équivalentes à celles qu'a supportées l'Allemagne ou l'ensemble de la zone euro. ces pertes sont restées à leur charge. Selon moi, cette situation découle du choix réalisé par le Gouvernement de recourir aux prêts garantis par l'État, plutôt qu'à des aides directes sur fonds publics. Il convient en revanche de souligner que les ménages dans leur ensemble- je dis bien dans leur ensemble, sans me prononcer sur des situations particulières, ni sur des catégories de populations pour lesquelles la précarité s'est accentuée -ont été préservés du choc économique, leur revenu brut ayant progressé. Au total, cette année d'exécution exceptionnelle du budget de l'État, mais aussi des comptes sociaux et des comptes des collectivités locales, s'accompagne d'une dégradation d'une ampleur inédite des comptes publics. Le solde des administrations de sécurité sociale et des administrations publiques locales devient déficitaire en 2020, tandis que le déficit budgétaire de l'État atteint le niveau inédit de 178 milliards d'euros. Je veux aussi souligner les conséquences très importantes des pertes de recettes tarifaires et domaniales subies par les collectivités territoriales, au-delà de la réduction de près de 2 % de leurs recettes issues des prélèvements obligatoires, et saluer la mise en oeuvre, puis la reconduction, de mécanismes de compensation adaptés, sous l'impulsion notamment de notre assemblée. En ce qui concerne l'emploi public,

Nous avons certes, dans un esprit de responsabilité, voté les quatre projets de loi de finances rectificative pour 2020, en obtenant d'ailleurs d'importantes évolutions, devenues des apports du Sénat. Nous avons en particulier adopté les mesures de soutien, essentielles pour maintenir les entreprises à flot et protéger les ménages. Toutefois, nous ne partagions pas les choix du Gouvernement qui ont guidé la construction de la loi de finances initiale pour 2020. En particulier, nous déplorions votre renoncement à redresser les comptes publics ; nous nous étions aussi opposés à de nombreuses mesures et avions regretté de n'avoir pas été entendus sur le schéma de financement des collectivités territoriales au titre de la suppression de la taxe d'habitation.

Au lieu d'être annulés, 36 milliards d'euros de crédits ont été reportés, et cela sans que la destination initialement prévue soit nécessairement respectée. Monsieur le ministre, cette pratique nuit au contrôle parlementaire. Elle est une entorse à la sincérité des lois de finances. Quoi qu'il en soit, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat de ne pas adopter ce projet de loi de règlement. J'en viens maintenant au débat d'orientation des finances publiques pour 2022. Dans mon intervention devant la commission, lundi dernier, j'ai principalement démontré que, une fois encore, cette étape de la procédure budgétaire n'apportait pas beaucoup plus d'informations que le programme de stabilité présenté en avril dernier. En effet, le rapport du Gouvernement, qui nous a été transmis le 30 juin, ne modifie pas la trajectoire des finances établie et confirmée par le programme de stabilité, puis le projet de loi de finances rectificative pour 2021, définitivement voté en début de semaine. En outre, le document ne permet pas vraiment non plus de lever le voile sur les intentions du Gouvernement pour les prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale. À peine constations-nous que les efforts pour redresser les comptes publics

je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, puisque, en réalité, c'était l'allocution du Président de la République qu'il fallait écouter ! En effet, lundi soir, le rapport préparatoire, transmis pourtant au Parlement une dizaine de jours plus tôt pour préparer notre débat,

Il est également permis de se demander si les mesures d'accompagnement de sortie de crise que nous venons de voter dans le cadre du projet de loi de finances rectificative suffiront vraiment, dès lors que la reprise de certaines activités pourrait se voir freinée par l'obligation de respecter le passe sanitaire, que ce soit dans les transports, les lieux de culture, l'hôtellerie-restauration ou

Par ailleurs, aucune révision des prévisions de croissance n'est opérée pour les années à venir. Pouvez-vous nous en dire davantage, monsieur le ministre ? Le Président de la République n'a pas uniquement révisé la croissance à la hausse il a également annoncé une série de dépenses supplémentaires, actuellement absentes de la trajectoire des finances publiques, à l'instar d'un plan d'investissement et d'un « revenu d'engagement » pour les jeunes sans emploi, dans le prolongement de la garantie jeunes universelle. Quel sera le montant de ce plan d'investissement ? Quel serait le montant d'un tel revenu garanti aux jeunes précaires ? Et comment seront-ils financés ? Autant de questions qui restent actuellement sans réponse, mais qui, à n'en pas douter, rendent obsolète le peu d'éléments qui figuraient dans le rapport du Gouvernement. ne disposons d'aucune information nouvelle sur la stratégie de redressement des comptes publics. Enfin, s'agissant du « tiré à part » sur les plafonds par mission et l'évolution prévisionnelle des emplois en vue du je note surtout un accroissement de près de 11 milliards d'euros des crédits du budget de l'État, qui n'inclut ni les appels en garantie ni les dépenses du plan de relance et du futur plan d'investissement. La plupart des missions du budget général sont concernées, sans que ces dépenses supplémentaires soient gagées par des économies, à l'exception d'économies de constatation sur le service public de l'énergie et de 150 millions d'euros au titre du plan d'économies sur les achats de l'État. Le « tiré à part » ne fait par ailleurs que confirmer votre renoncement à la baisse de l'emploi public,

au service du redressement et de l'amélioration de nos indicateurs budgétaires et fiscaux. Nous en reparlerons cet automne, mais les échanges de ce jour s'en trouvent amputés d'autant, ce qui ne sert pas le débat parlementaire auquel nous sommes pourtant tous très attachés. La parole

c'est la première fois que je m'exprime devant vous en tant que rapporteure générale de la commission des affaires sociales. En cet instant, je souhaite tout d'abord redire ma gratitude envers mon prédécesseur, Jean-Marie Vanlerenberghe, qui a su, durant sept ans, défendre avec constance l'action de la sécurité sociale et de ses différentes branches et plaider pour la gestion rigoureuse de ses comptes, au nom de la soutenabilité et de la pérennité de notre modèle social. Pour en venir au fond, au moment où il m'incombe de reprendre ce flambeau, la situation des comptes sociaux est particulièrement préoccupante. Elle l'est dans l'immédiat. Vous l'avez souligné, monsieur le ministre, la sécurité sociale a enregistré en 2020 le plus lourd déficit de son histoire, et de loin : 38,7 milliards d'euros sur le périmètre du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse, et même 39,8 milliards d'euros si on l'élargit à l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Cela fait environ 10 milliards d'euros de plus que le précédent record, qui datait de 2010, au plus fort de la crise financière entamée en 2008. Pour 2021, selon les dernières prévisions de la commission des comptes de la sécurité sociale, le déficit du régime général et du FSV devrait rester stable à environ 38,4 milliards d'euros, malgré des recettes nettement plus élevées que prévu. au-delà de cette photographie de crise, la situation des comptes sociaux est préoccupante à moyen terme. La trajectoire financière pour les quatre prochaines années, annexée à la dernière loi de financement de la sécurité Ainsi, selon les projections du Gouvernement, le déficit se stabiliserait à près de 20 milliards d'euros à l'horizon 2024, soit un niveau très élevé, voire vertigineux. Or ce n'est pas en regardant dans le rétroviseur que nous pourrons nous rassurer. En effet, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas parvenus à ramener les comptes de la sécurité sociale dans le vert avant la crise sanitaire, une décennie après la crise financière de la fin des années 2000, en partie, monsieur le ministre, parce que le Gouvernement n'a pas souhaité cet excédent et l'a assumé au travers de diverses mesures de non-compensation. Certes, être dans le rouge, et même dans le rouge vif, ne distingue pas les comptes sociaux de ceux des autres administrations publiques, en particulier de ceux de l'État. Mais il me semble important de rappeler la spécificité des comptes sociaux au sein de l'ensemble des comptes publics, car cette spécificité semble parfois oubliée dans certains ministères au profit de formules faciles se référant à « la même poche ». Les dépenses de la sécurité sociale, de même que celle des autres régimes d'assurance sociale obligatoires, sont fondamentalement des dépenses de répartition. Des prestations sociales sont versées à partir des produits collectés, c'est-à-dire encore majoritairement des cotisations créatrices de droit et fléchées à cette fin vers un organisme précis. À l'inverse des dépenses de l'État, il n'y a que très peu de dépenses d'investissement ou même de dépenses d'avenir, comme pour l'éducation, l'enseignement supérieur ou la recherche,

Au contraire, il devrait être de la responsabilité de chaque génération d'assurer elle-même le coût de sa protection sociale, bref de ne pas faire payer à ses enfants le prix de ses feuilles de soins ou des actuelles retraites, par exemple. C'est donc bien la recherche de l'équilibre, au sens strict du terme, qui doit nous guider quand on parle des comptes sociaux. C'est d'ailleurs ce constat qui a amené votre prédécesseur Jean Arthuis à mettre en place

Monsieur le ministre, Jean-Marie Vanlerenberghe vous avait dit l'année dernière, lors de l'examen des projets de loi relatifs à la dette sociale et à l'autonomie, que, face à l'ampleur des conséquences financières de la crise sanitaire, nous étions en quelque sorte revenus au point de départ en matière de dette sociale, vingt-cinq ans après. Il était donc temps de se poser de nouveau les questions fondamentales nous donnons-nous vraiment pour but d'éteindre la dette sociale, dans l'esprit de responsabilité vis-à-vis des générations futures dont je viens

Dès lors, nous devons nous montrer cohérents et réellement agir pour atteindre cet objectif. Cela commence par ne pas priver artificiellement la sécurité sociale de ses recettes, par ne pas lui confier par commodité des charges qui étaient jusqu'en 2019 celles de l'État- je pense à Santé publique France, par exemple -et par ne pas faire de la Cades un « fourre-tout », par exemple en la chargeant à hauteur de 13 milliards d'euros du financement des investissements des hôpitaux publics. Sinon, monsieur le ministre, nous n'y arriverons pas, et autant supprimer tout de suite la Cades Bien sûr, le respect de ces principes élémentaires de bonne gestion des finances publiques ne suffira pas, à lui seul, à ramener les comptes de la sécurité sociale sur le chemin de l'équilibre. Soyons conscients, mes chers collègues, qu'il faudra prendre, le moment venu, à l'issue de la crise actuelle, des décisions difficiles, notamment en matière d'assurance vieillesse ou de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Pour nous y aider, et afin que le Parlement dispose des moyens d'exercer pleinement les prérogatives qui devraient être les siennes en matière de finances sociales, nous formulerons des propositions cet automne, dès l'examen de la révision du cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale. À cet égard, je vous rappelle les principes sur lesquels s'appuie la proposition de loi organique déposée par Jean-Marie Vanlerenberghe et notre présidente Catherine Deroche,

dont la situation financière et le niveau d'endettement sont très préoccupants. Ensuite, elle instaure une normativité renforcée, en particulier par la mise en place de certains crédits limitatifs,

sur le modèle de la loi de règlement que le Sénat va examiner à l'issue de ce débat. Enfin, le texte met en place une « règle d'or »- nous en avions discuté l'année dernière -imposant un équilibre des comptes de la sécurité sociale sur cinq années glissantes, sur le modèle de ce qui était prévu pour le système universel de retraite. Si les modalités et la date de mise en place d'une telle règle peuvent bien sûr être discutées, son principe devrait nous unir, pour peu que nous fondions notre jugement sur nos échecs passés.

le moment est enfin venu de clore l'exercice budgétaire 2020. Cette année, qui restera dans l'histoire comme celle de la grande dépression sanitaire, aura profondément éprouvé notre économie et nos finances publiques. Nous ne sommes pas près d'en oublier les chiffres record : un déficit public qui est passé au-delà de 9 % du PIB, un endettement public qui a bondi de 18 points en moins d'un an, une dépense publique qui a franchi les 60 % du PIB. Il est grand temps de tourner la page de ces tristes records budgétaires. Pourtant, quel que soit le sort que le Sénat réservera à ce texte, il nous faudra bien- je m'adresse à chacun d'entre vous, mes chers collègues -assumer les conséquences des mesures sanitaires que nous avons prises pour protéger le pays. c'est bien là tout l'enjeu de nos discussions de cette après-midi : dans quelle mesure sommes-nous disposés à assumer les conséquences économiques et politiques de Je le répète, cette question va bien au-delà de considérations strictement budgétaires, considérations auxquelles le projet de loi de règlement nous invite pourtant. En effet, notre assemblée a déjà tranché le sort des quelque 70 milliards d'euros de mesures d'urgence. La majorité du Sénat a voté les quatre projets de loi de finances rectificative pour 2020. Chaque fois, une solution de compromis a été trouvée, soit dès la première lecture, en mars 2020, soit lors de la réunion de la commission mixte paritaire, pour les trois textes suivants. Chaque fois, la chambre haute a accepté, directement ou indirectement, les dérapages contrôlés qui nous éloignaient un peu plus de la trajectoire retenue dans la loi de finances initiale, au point de laisser les critères de Maastricht, sur le déficit comme sur la dette, à des années budgétaires de notre portée.

S'agissant du programme 231, « Vie étudiante », les crédits de paiement inscrits dans le projet de loi de règlement sont ainsi supérieurs de 8,5 % à ceux qui figuraient en loi de finances initiale. Les subsides versés aux étudiants pour les aider à surmonter la crise sanitaire ont causé une augmentation des dépenses de 166 millions d'euros pour la seule année 2020. Il en va de même pour le « plan Étudiants », dont le budget s'est également envolé. Comme j'ai eu l'occasion de le préciser dans mon rapport, nous pouvons regretter que ces dépenses supplémentaires viennent s'ajouter à des lignes de crédits qui méritaient déjà, avant la crise, une évaluation rigoureuse. J'ai parlé de la mission « Recherche et enseignement supérieur », mais ce constat vaut aussi pour toutes les autres missions. Cette mission revêt toutefois, reconnaissons-le, mes chers collègues, une valeur symbolique bien particulière, car elle concerne des dépenses que nous avons décidé d'engager au bénéfice exclusif des jeunes générations. Or c'est naturellement sur elles que nous comptons pour rembourser les dettes que nous contractons aujourd'hui. Tel est le contrat que nous avons passé avec les jeunes générations. C'est l'esprit de responsabilité qui nous oblige, c'est aussi notre intérêt collectif, car nous nous attachons ainsi à soigner, tant que nous le pouvons encore, la signature de la France sur les marchés financiers. C'est le meilleur moyen dont nous disposons pour préserver notre capacité à emprunter, donc à financer nos propres projets.

Nous serons ainsi en cohérence avec nos décisions passées et nous aurons un cap pour l'avenir. S'agissant de ce cap, nous aurons l'occasion dès l'automne d'affirmer nos positions et d'avancer des propositions concrètes d'orientation des finances publiques. Pour nous, la priorité demeure la réduction de l'endettement public. Il y va de notre capacité collective à investir dans la nécessaire réindustrialisation, notamment par la redynamisation des chaînes de valeur, et dans les technologies du futur, à accélérer la transition écologique, à préserver notre modèle social. Bref, il y va de notre souveraineté nationale.

Il y a l'ampleur de ces reports de crédits de 2020 vers 2021- ils représentent une trentaine de milliards d'euros. Vous plaidez la prudence ... C'est bien, mais notre interrogation sur la sincérité budgétaire et la portée réelle de l'autorisation parlementaire est plus ample que cela. Nous avons souvent alerté sur l'illisibilité de la répartition des crédits entre ce qui relevait de l'urgence, de la relance et du budget ordinaire. S'y ajoute la question des comptes sociaux. À force de prélèvements et de remboursements, d'exonérations de cotisations, l'autonomie de la sphère sociale est aujourd'hui une chimère. L'État décide, la sécurité sociale paie, et les flux financiers entre les deux sont de plus en plus insaisissables.

ou versant des dividendes soit bénéficiaire du fonds de solidarité ou des aides du plan de relance, alors que, en même temps, l'État a renforcé les contrôles sur les Français ? J'en veux pour preuve cette réforme de l'assurance chômage, qui

le résultat ! Nous sommes face à une gestion de crise profondément déséquilibrée, avec, d'un côté, une crise sociale minimisée, de l'autre, une richesse indécente qui s'étale dans les colonnes des journaux. Le magazine a publié, la semaine dernière, son classement annuel des fortunes du pays et constate, je cite, « les plus fortes progressions annuelles jamais enregistrées ».

l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, ses efforts pour rénover l'économie américaine, en commençant par les infrastructures, la transition écologique et la consommation populaire. Je citerai les discussions mondiales, freinées par la France-

Alors, oui, vous mettez de l'argent public sur la table, mais c'est à notre tour de vous demander de ne pas faire de dépenses dans le vide ou sans résultat ! Pendant des années, nous, les écologistes, la gauche, avons demandé des moyens

aux 90 milliards d'euros de dépenses fiscales, pour une grande partie « brunes » et finançant les pollutions. Il faut conditionner toutes les aides d'État à des critères sociaux et environnementaux et évaluer la performance des milliards d'euros Cette crise a réhabilité l'État. C'est une grande victoire. Mais notre appareil d'État a été abîmé par des décennies de coupes, de management néolibéral, de pertes de compétences et d'externalisations. Voilà le combat des prochaines années, pour nous qui devons contrôler les autorisations budgétaires et les finances publiques s'assurer que l'État soit en capacité de faire bon usage des crédits que nous votons. Il faudra, par exemple, s'interroger sur l'ampleur de l'argent public dépensé en audits et prestations de sociétés de conseil pour pallier la perte de compétences en interne. On l'a bien vu au coeur de la crise, lorsque des cabinets privés

la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en toute responsabilité et avec l'envie de préserver notre pays des effets de la crise que nous avons adopté les quatre projets de loi de finances rectificatives pour 2020 dès la première lecture, ces textes ayant reçu un large soutien sur ces travées.

vous, qui ont voté à nos côtés tous les PLFR, choisissent de s'abstenir ou de rejeter ce texte. Certains l'ont déjà dit, ce projet de loi de règlement s'illustre, à la fois, par un écart important avec la loi de finances initiale et par d'importants reports de crédits. L'écart à la loi de finances initiale n'est pas surprenant au regard des montants que je viens d'évoquer et des quatre PLFR que la crise nous a contraints d'adopter. Les quelques « surbudgétisations », qu'il est bien facile de constater, de constater, me semblent témoigner uniquement de la prévoyance du Gouvernement. Certes, elles concernent des montants importants, mais n'oublions pas trop vite le contexte d'incertitude dans lequel les PLFR ont été adoptés. Qu'auriez-vous dit si le Gouvernement, s'appuyant sur des hypothèses trop optimistes, n'avait pas prévu des enveloppes assez larges pour financer les mesures d'urgence ?

Bien entendu, nous en voyons la traduction directe dans la loi de règlement, avec d'importantes enveloppes de crédits non consommés en 2020, crédits dont le report nous a d'ailleurs permis d'affronter les nouvelles restrictions intervenues en avril dernier. Comme vous tous, mes chers collègues, je suis attaché à l'esprit de la LOLF, à la sincérité et à la bonne tenue de nos comptes publics. Mais soyons honnêtes, cette sous-consommation est une bonne nouvelle pour nos comptes publics. Elle est le signe de la prévoyance du Gouvernement, et je la crois inévitable en période de crise. Venons-en maintenant à la question du déficit et de la dette. Là encore, c'est une situation qui nous préoccupe tous, et la sortie de crise devra être l'occasion de veiller à rétablir l'équilibre de nos finances.

ne faisons pas de ce vote un prétexte ! J'ose espérer que ceux d'entre vous qui ont voté, à nos côtés, chacun des PLFR de 2020 sauront s'en souvenir et auront le courage d'en tirer les conséquences par leur vote de ce jour. ailleurs, le temps approche où nous pourrons discuter en profondeur de nos règles budgétaires et de la transformation du pilotage des finances publiques. La proposition de loi de nos collègues députés Éric Woerth et Laurent Saint-Martin est une première étape. Il faudra nous saisir au-delà des clivages partisans ou de nos désaccords du moment : pour les générations futures, il est dans l'intérêt de tous d'améliorer la gestion de nos finances publiques. Mais comment ? Comment agir pour rééquilibrer les finances publiques sans recourir à des hausses d'impôts, alors que la dépense publique ne cesse d'augmenter depuis plus de cinquante ans ? Mes chers collègues, le temps est venu de se doter de nouveaux outils, qui nous permettront de transformer efficacement et rapidement notre gouvernance financière. La commission présidée par Jean Arthuis a proposé trois pistes en ce sens à chaque nouvelle mandature, nous pourrions voter une norme de dépense pluriannuelle qui fixerait une trajectoire à respecter ; nous pourrions doter la France d'une nouvelle institution indépendante chargée d'évaluer l'impact des politiques publiques sur nos finances et de faire des prévisions macroéconomiques à plus long terme renforcer les temps de contrôle de l'exécution budgétaire pour l'ensemble des administrations publiques et instituer une loi de règlement pour le PLFSS. Mes chers collègues, être l'occasion de trouver des solutions nous permettant d'accompagner les réformes structurelles qu'a rappelées le Président de la République et de rénover la gestion de nos finances publiques avec lucidité et ambition.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, madame, monsieur les rapporteurs généraux, mes chers collègues, comme il est d'usage chaque année, nous consacrons une séance conjointe à l'examen du règlement du budget de l'année précédente et au débat d'orientation en vue du budget de l'année suivante. Le Sénat a l'habitude de cet exercice d'équilibriste entre passé, présent et avenir. Le temps limité et le placement en fin de session extraordinaire font que ces

J'en viens au projet de loi de règlement de 2020. Sur le fond, il apparaît difficile, si nous voulons être cohérents, de voter contre un budget dont nous avons globalement approuvé les nombreuses révisions l'an dernier. Il s'agit en quelque sorte de l'équivalent, pour l'État, du compte administratif qui doit être voté dans nos collectivités avant le 30 juin. Ce vote devrait donc être un vote de cohérence sur un texte constatant l'exécution budgétaire, même si l'on peut regretter des « incidents », comme les importants reports de crédits sur 2021. La situation est moins nette pour le présent et l'avenir. La prévision de croissance économique du Gouvernement, dans le programme de stabilité du printemps et dans le budget 2021 révisé, s'établit à 5 %. Mais selon la plupart des instituts de prévision, elle se situerait plutôt entre 5,5 % et 6 %. Dans son allocution de lundi dernier, le Président de la République semble avoir corroboré cette hypothèse, en parlant d'une croissance à 6 % en 2021. Ces hypothèses restent très dépendantes de l'évolution de la situation, en particulier sanitaire, cet été et à l'automne ... Disons que les prévisions actuelles pour 2021 et 2022 nous permettent d'espérer un rattrapage du choc historique dans environ deux ans. en va autrement du retour à l'équilibre budgétaire. Le Gouvernement annonce un « effort de consolidation » à partir de 2023. Le retour en dessous des 3 % de déficit, lui, n'interviendrait pas avant 2027, soit la fin du prochain quinquennat. Je pense également au budget de la sécurité sociale, durement affecté par la crise sanitaire. Pour y parvenir, le montant des économies à réaliser se chiffre en dizaines de milliards d'euros, alors même que nous devrons réaliser des investissements massifs dans la transition énergétique et que nous souhaitons maintenir un degré acceptable de solidarité. Cette législature porte la responsabilité du surcroît exceptionnel d'endettement public contracté sur Toutefois, la hausse de l'endettement public depuis trente ans est une responsabilité politique collective. Il est donc vain de vouloir attribuer à tel ou tel camp politique l'entière responsabilité de cette situation. Même si trop peu a été fait avant la crise sanitaire, et trop lentement, nous devons reconnaître que la réduction du déficit public avait été continue pendant près de dix ans. L'actuelle majorité avait d'abord affiché des objectifs ambitieux en la matière, malgré la difficulté, bien connue, de toute gestion des finances publiques. Pour la première fois depuis dix ans, le solde était repassé en 2018 sous le seuil de 3 % de déficit. On peut saluer un réel effort de « sincérisation » du budget et des hypothèses globalement raisonnables avant 2020, malgré une réduction trop timide du déficit structurel. À moyen terme, le Gouvernement prévoit une stabilisation de la dette publique autour de 118 % du PIB. Pour cela, on entrevoit déjà la poursuite des réformes structurelles. Peut-être faudrait-il aussi tabler sur des solutions moins « orthodoxes », comme un retour de l'inflation En conclusion, les membres du RDSE voteront majoritairement pour l'adoption du projet de loi de règlement et expriment des attentes fortes en vue de la présentation du budget pour 2022 à la rentrée, en termes tant de bonnes recettes que de bonnes dépenses.

et de tenir compte de la reprise épidémique à laquelle nous faisons face ». Vous n'aviez pas besoin de cet argent, puisque 31,6 milliards d'euros n'ont pas été dépensés ! La Cour des comptes évoque un « manque de réalisme des prévisions budgétaires ». La ficelle est grosse Vous avez reporté un montant de crédits inégalé, qui représente onze fois plus que le maximum observé lors de ces dix dernières années. Il fallait vous croire sur parole, alors même que les faits vous trahissent depuis 2017

à 32 % chez les jeunes, et la situation est pire pour les indépendants. Les pauvres sont encore plus pauvres. Le maintien des recettes de l'impôt sur le revenu pour l'année n'y change rien- la moitié des Français ne le paie pas -, et, pour les autres, l'actualisation de leur taux entraînera des remboursements d'impôts causés par leur appauvrissement. Parlons du décret d'avance de 7,2 milliards d'euros. Nous sommes loin du temps où le candidat Macron se prévalait du « sérieux budgétaire pour ne pas léguer une dette insoutenable à nos enfants ». Le candidat, devenu Président de la République, fait voter par son gouvernement un budget déficitaire de 84,9 milliards d'euros,

Alors que la centaine de milliardaires français voit sa fortune augmenter de 300 milliards d'euros pendant la crise, le Gouvernement, tout comme la majorité sénatoriale, se refuse à trouver de nouvelles recettes.

République a parlé, le Gouvernement acquiescera et le Parlement validera. Et voilà ! Le budget serait déjà arrêté sur un plateau de télévision lors d'une allocution présidentielle. d'une intervention culpabilisante pour la majorité des Français, qui organise ce que j'appelle le désordre dans les institutions publiques, dans le secteur privé comme dans le secteur public, dans le quotidien des Français. Le choix est clair : orchestrer la concurrence violente entre les individus et octroyer toujours plus de dispenses au capital. La réforme de l'assurance chômage sera appliquée dès octobre prochain, une marque d'obstination contradictoire avec la prétendue mobilisation pour les salariés des entreprises n'ayant pas résisté à la crise.

Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a lui aussi contredit les velléités du président-candidat de détruire le système de retraite, quitte à inventer des problèmes qui n'existent pas. Ainsi, d'après le COR, « malgré le contexte de la crise sanitaire et le vieillissement progressif de la population

Le Parlement, le Conseil d'État, les syndicats, le peuple ... Ce sont des détails ! Le désordre organisé frappe le déroulement de nos débats. Nous n'échangeons plus que sur des décisions déjà arrêtées.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour la deuxième année consécutive, il nous est présenté un projet de loi de règlement des comptes de l'État dans des circonstances exceptionnelles, avec des conditions sanitaires économiques et sociales dégradées. dégradées. Cet examen est l'occasion, pour mon groupe, de revenir sur les choix budgétaires qui ont été les vôtres durant cette année. La politique du « quoi qu'il en coûte », qui a bien entendu pesé sur les comptes publics, n'est évidemment pas remise en question, question, alors même que le « quoi qu'il en coûte » va coûter très cher aux mêmes. Je salue au passage la volonté du Gouvernement de faire passer en force, coûte que coûte, un dérivatif de réforme des retraites- elle n'est ni faite, ni à faire -, ainsi que la réforme de l'assurance chômage, qui arrive à point nommé alors que la France compte 8 % de chômeurs. En revanche, il est des fondamentaux intangibles dans vos politiques budgétaires. Tout d'abord, monsieur le ministre, en conduisant une politique de l'offre et en « oubliant », contre l'avis de la très grande majorité des économistes, toute politique de la demande, vous laissez se creuser les inégalités et se développer la pauvreté, après un début de quinquennat pourtant très marqué par les dégâts causés en la matière. Vous aviez déjà casé dans le plan de relance

Ces choix-là sont tout sauf neutres ; ils portent en eux, l'idéologie qui vous anime en la matière. En effet, cela fait près de vingt-cinq ans qu'une telle politique est suivie de très peu, voire d'aucun effet sur l'emploi et la compétitivité. de manière significative la protection sociale de recettes. Ironie du calendrier, l'Insee vient de souligner combien la protection sociale était essentielle face à la tendance du capitalisme français à l'augmentation des inégalités de revenus primaires les 20 % les plus aisés empochent neuf fois ce que gagnent les 20 % les plus pauvres. C'était sept fois en 2008 ... De plus, votre politique budgétaire en matière d'aides souffre d'un manque cruel de conditionnalité de ces dernières, particulièrement vis-à-vis des grands groupes. Un récent rapport de l'Observatoire des multinationales a pourtant montré que, sur les 27 groupes du CAC 40 qui ont bénéficié de l'activité partielle, 16 ont versé des dividendes en 2020 et 22 en 2021. manifestement pas assez d'argent pour faire travailler les salariés à plein temps, car il faut rémunérer les actionnaires ! En pleine pandémie, les entreprises du CAC 40 distribuent ainsi en dividendes l'équivalent de 140 % de leurs profits. Elles ont dû prendre dans leur trésorerie ou s'endetter pour cela.

Enfin, comme le diagnostiquait l'Institut Montaigne dès décembre dernier, il manque 30 milliards d'euros d'aides, celles qui devraient aller vers les plus démunis que sont les chômeurs, les jeunes et les familles monoparentales.

Non seulement votre gouvernement ne veut pas aider les pauvres, mais en plus il leur retire de l'argent. Et, de grâce, ne nous dites pas que « l'argent magique » n'existe pas

Je rappelle que cet impôt a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, qui rapportait environ 4 milliards d'euros. Inutile d'être haut fonctionnaire à Bercy pour comprendre que près de 2,5 milliards d'euros se sont perdus en route

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment d'examiner l'exécution des autorisations d'engagement et des crédits de paiements prévus par le projet de loi de finances pour 2020, il n'est pas inutile de rappeler la responsabilité du Gouvernement dans une guerre sanitaire qu'il a été incapable d'anticiper et de maîtriser et qui aura coûté à notre pays, en plus d'« un pognon de dingue », la perte inestimable de 111 000 vies. Il n'est pas inutile de rappeler que les recettes nettes de l'État ont diminué de 33 milliards d'euros, tandis que les dépenses ont augmenté de 46 milliards d'euros par rapport aux prévisions budgétaires légales. La dette s'établit à près de 116 % du PIB à la fin de 2020, tandis que le déficit public atteint 178 milliards d'euros. Dire, monsieur le ministre, que vous avez le toupet de nous faire la leçon sur la compétence de votre gestion ! Votre incompétence, globale, je l'illustrerai par deux missions qui me tiennent à coeur. La première est Malgré une baisse exceptionnelle de 40 % des demandes d'asile, les dépenses liées ont été supérieures à ce qui était prévu dans le PLF pour 2020. Il n'y a manifestement aucune maîtrise des dépenses sur ce point. De plus, le ministère de l'intérieur refuse encore et toujours de communiquer le coût de l'immigration pour nos collectivités territoriales et nos services de protection sociale, alors que ces données devraient être annexées au projet de loi de finances ou au projet de loi de règlement. C'est un impératif de transparence. Mais, de Beauvau à Bercy, on préfère taire la réalité Il ne faut absolument pas que les Français sachent que, en plus d'être un fléau pour notre identité, notre sécurité et notre économie, l'immigration est une calamité pour nos comptes publics. Quant à l'aide au développement- la seconde mission -, qui n'est rien d'autre que l'aide publique française accordée au développement des pays étrangers, elle atteint près de 13 milliards d'euros cette année. De nombreuses dépenses humanitaires d'État ont été surexécutées en 2020. La dette du Soudan se voit ainsi généreusement allégée de 4 milliards d'euros, pendant que Bercy exige de nos TPE et PME le remboursement du prêt garanti par l'État. cette générosité, d'un côté, et de cette haine de soi, de l'autre, est une spécialité française et une forme de naïveté économiquement suicidaire. Aussi, plutôt que de faire plus pour l'Afrique, il est impératif de faire plus pour la France. Elle est là, la véritable justice sociale Pour les orientations budgétaires, je propose donc de rattraper la calamiteuse gestion de la crise sanitaire sans augmenter les impôts, mais en luttant contre la fraude sociale, qui s'élève à 20 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes et à 50 milliards d'euros selon le magistrat spécialiste Charles Prats. combattre la fraude fiscale, qui prive l'État et les collectivités locales de 80 milliards d'euros de recettes par an. Je propose d'en finir avec la folie migratoire, illégale ou légale, qui plonge notre pays dans le chaos fiscal. d'exiger de notre geôlier européen qu'il rende l'argent que vous et vos prédécesseurs avez consenti à lui transférer et qui nous prive de 7 milliards d'euros d'investissements chaque année. Je m'oppose donc au « quoi qu'il en coûte » planétaire et autoritaire, pour instaurer une légitime priorité, voire exclusivité, nationale, sociale et démocratique. Les 10 millions de pauvres que compte notre pays l'exigent, monsieur le ministre. Du cadre feutré de nos débats, sortons nos esprits confinés : plutôt que de culpabiliser et de diviser les Français, sachez enfin les rassembler, les réconcilier et les protéger

de restrictions réglementaires importantes dans les services et de charges administratives significatives, de même que des niveaux et une efficacité faibles des investissements dans la

nous avons diminué en relatif nos actions dans les domaines de la défense, de la famille, de l'enseignement et de la santé ; dans le même temps, nous avons augmenté nos dépenses pour le chômage et les retraites.

le rapport note une stabilité des effectifs de l'État et de ses opérateurs, avec un renforcement des moyens dans la police et dans la justice, qui sera contrebalancé par une réduction dans tous les secteurs où cela est possible. On a l'objectif, mais pas les moyens

de répondre à une absence de crédits budgétaires. Je ne citerai qu'un seul exemple : le plan Nano 2022. Sur les réformes structurelles, la Cour des comptes relève que la croissance économique est une condition nécessaire au redressement de nos finances publiques, tout en précisant qu'elle n'est pas une condition suffisante pour une décrue durable de notre dette. Comme cela a été dit, il faut agir sur la dépense et surtout améliorer son efficacité. La France a creusé son écart avec ses partenaires européens « sans que les indicateurs économiques, sociaux, de développement humain ou en termes de qualité

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, encore une fois, je salue la qualité du service de la communication de Bercy.

Avant la gestion de la crise sanitaire, notre situation budgétaire était très mauvaise ; contrairement à vous, monsieur le ministre, je ne vois pas où étaient les marges budgétaires. Au demeurant, après la gestion de la crise, elle est extrêmement mauvaise.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 est indéniablement singulier. En effet, il vient clore les comptes d'une année marquée par la plus grave crise que nous ayons eu à traverser depuis la Seconde Guerre mondiale. Fait inédit dans l'histoire budgétaire de notre pays, pas moins de quatre lois de finances rectificatives ont dû être votées par le Parlement pour définir, ajuster, puis recharger les différents mécanismes de soutien à la vie économique du pays. Contre le cataclysme économique provoqué par la propagation du virus et la suppression d'une partie substantielle de l'offre productive, l'État a pris des décisions inédites, en ouvrant grand les vannes de la dépense publique. À l'effet de ces mesures de soutien s'est ajouté celui de la contraction de l'activité économique sur l'encaissement des recettes publiques. Résultat : la France a vu son déficit public se dégrader de plus de 137 milliards d'euros- vertigineux ! -, et ce pour répondre dans l'urgence à la déflagration de la situation liée au covid-19 et atténuer l'impact des conséquences économiques et sociales de la crise aussi bien sur les familles et les entreprises que sur les collectivités locales. Le déploiement des mesures d'urgence était nécessaire ; à une écrasante majorité, et sur toutes les travées, nous les avons largement soutenues. Les soutiens publics au titre du chômage partiel ou du fonds de solidarité relevaient d'un impératif de sauvegarde du tissu économique et social.

du principe de sincérité, comme marque de l'exécutif dans la gestion des comptes publics. Or le dévissage de nos comptes publics traduit surtout le manque d'anticipation et d'efforts du Gouvernement en matière d'assainissement des comptes publics. Oui, si la France avait eu des finances publiques plus saines au début de l'épidémie de covid-19, nos marges de manoeuvre auraient été plus grandes aujourd'hui. L'absence de réformes structurelles passées est donc un handicap non seulement pour le temps présent, Si l'État est légitime à s'endetter, en particulier en période de relance économique, il ne peut pérenniser un haut niveau d'endettement sans sacrifier notre prospérité de demain, celle de nos enfants. C'est d'ailleurs ce qui nous avait motivés à rejeter, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2020.

Place au volontarisme, afin d'assainir les comptes de la Nation ! En ce sens, le choix du Gouvernement de ne pas imputer au solde structurel les mesures liées à la crise sanitaire ne fait que renforcer l'illisibilité de la stratégie des finances publiques pour les années à venir. En bref, le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 est le reflet d'une situation exceptionnelle pour laquelle un effort budgétaire immédiat était indispensable. À moyen terme, la relance économique doit porter ses fruits. À long terme, nous ne pourrons faire l'économie d'une véritable stratégie de redressement des comptes publics, afin de conserver la maîtrise de nos finances publiques, en direction des collectivités locales.

paix, a rendu dérisoires les efforts budgétaires opérés au début du quinquennat en faveur des finances publiques, car les sacrifices sur lequel ils reposaient sont douloureux. J'en donnerai deux exemples : la chute de la production de logements depuis le début de ce quinquennat- on sait à quel point cela pèse sur le pouvoir d'achat des Français -et la

On peut et l'on doit maîtriser les finances publiques avec la volonté de réduire les inégalités, avec le souci de l'équilibre et de la justice, avec le souci de la capacité d'action publique. C'est d'autant plus essentiel après cette crise

Même la suppression de la taxe d'habitation, maintenue en 2022-2023, va accroître les inégalités, alors que, dans le programme du candidat Emmanuel Macron, elle était présentée comme une mesure de lutte contre les inégalités.

des « gilets jaunes ». Je remarque que, à défaut de se réinventer, le Gouvernement est aujourd'hui sur la défensive. Il reconnaît que sa politique n'est plus adaptée, puisqu'il renonce aux baisses d'effectifs prévues dans la fonction publique. Je me réjouis de ce renoncement, publique. Je me réjouis de ce renoncement, mais un renoncement ne fait pas une politique. Quelles sont donc les perspectives du Gouvernement à l'heure actuelle ? L'extinction la plus rapide possible des mesures de soutien ? Restons prudents. La réforme des retraites ? On ne sait plus trop laquelle. La réforme de l'assurance chômage, sans cesse reportée, tellement elle est douloureuse ? Pendant ce temps, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a augmenté de 30 %. Pour nous, il n'est pas possible de parler de l'avenir des finances publiques sans lier cette question aux deux grands enjeux de l'avenir : la transition écologique et la lutte contre les inégalités.

La crise économique la plus grave que nous ayons connue après la Seconde Guerre mondiale a entraîné mécaniquement une dégradation de nos finances publiques, à un niveau jamais atteint depuis 1944 chute des recettes fiscales, hausse massive des dépenses d'urgence et de relance pour sauver notre économie et, par voie de conséquence, niveaux de déficit et de dette publique record.

résulte de l'absence d'efforts suffisants de redressement de nos comptes publics au début du quinquennat. Selon le rapport préparatoire du Gouvernement au présent débat, « l'effort de maîtrise des comptes publics opéré de 2017 à 2019 a permis de disposer de marges de manoeuvre pour répondre de manière efficace

Notre déficit public avant-crise était de - 3,1 % en 2019 ; il était, avec celui de la Roumanie, le plus important des vingt-sept États membres de l'Union européenne. Les deux tiers des États membres étaient alors en excédent budgétaire et la moyenne des comptes publics en Europe était à l'équilibre. Nous ne disposions donc d'aucune marge de manoeuvre budgétaire pour financer les mesures de sauvegarde de notre économie, contrairement à la plupart de nos voisins européens, à commencer par l'Allemagne, qui disposait de plus de 13 milliards d'euros d'excédent budgétaire. Si notre groupe se félicite que les impôts n'aient pas été augmentés, il déplore toutefois l'absence d'économies au début du quinquennat. Exactement comme sous le quinquennat précédent, les économies n'ont cessé d'être repoussées à plus tard : réforme des retraites continuellement reportée, abandon de la promesse de réduction de 50 000 emplois au sein de l'État et de ses opérateurs. Comme l'a souligné la Cour des comptes en 2019, les dépenses publiques françaises étaient les plus élevées de l'Union européenne, se situant 8,8 points au-dessus de la moyenne, sans pour autant montrer toute leur efficacité.

haut. Comme le remarquait encore récemment Jean Peyrelevade, notre attractivité continuera d'être interrogée et la question des fonds propres des entreprises, que j'ai déjà évoquée ici, est devant nous. Résultat : alors que la France et l'Allemagne avaient le même niveau de dette avant la crise de 2008, un écart de 40 points s'est creusé entre elles en 2019.

locales. Selon la Cour des comptes, en 2020, l'épargne brute globale des collectivités locales a diminué de plus de 10 % et les dépenses d'investissements se sont contractées de 7,1 %. Certaines communes ont été particulièrement touchées.

2020 ? des conséquences importantes en matière de potentiel fiscal, donc de péréquation, liées à la réforme de la taxe d'habitation ? Le dispositif de neutralisation des indicateurs financiers qui servent à la répartition des dotations et des fonds de péréquation sera-t-il reconduit en 2022 ? en 2022 ? Attention à ne pas faire payer demain la note de la crise aux collectivités, comme on commence à le lire ici ou là ! Cette piste figurait dans le rapport de Jean Arthuis sur l'avenir des finances publiques et on la retrouve dans le projet de loi d'orientation des finances publiques. publiques. Les collectivités territoriales ne sont en rien responsables de ce déficit. Elles n'empruntent que pour investir et ne concourent qu'à hauteur de 2 % à la dégradation du solde public. En conclusion, si nous avons soutenu le Gouvernement dans la lutte contre la crise économique en 2020, nous n'avons pas cautionné l'état des comptes publics du début d'année, avant la survenance de cette crise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons modifié le projet de loi de finances initiale pour 2020.

pense notamment aux crédits du programme 203 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur spécial : les 4 milliards d'euros de recapitalisation de la SNCF ont été intégralement reportés, alors même que la situation financière

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, madame, monsieur les rapporteurs généraux, mes chers collègues, nous débattons cet après-midi tout à la fois du projet de loi de règlement de l'année passée et de l'orientation de nos finances publiques pour 2022. Si la jonction de ces deux sujets est naturelle pour que l'examen du passé éclaire les décisions à venir, l'exercice paraît frustrant à plusieurs titres.

L'exercice 2020 a été marqué par de nombreux collectifs budgétaires en cours d'année, destinés à ouvrir les crédits rendus nécessaires pour soutenir les entreprises et les ménages, et par une très forte dégradation de nos comptes publics. Si le Sénat a souscrit aux ouvertures de crédits, certains d'entre nous- et j'en fais partie -auraient souhaité des arbitrages différents, notamment en direction des jeunes et des publics les plus fragilisés par la crise. Par ailleurs, je suis de ceux qui pensent que, tout particulièrement en année de crise, alors que notre déficit public se creusait toujours davantage, les baisses d'imposition non ciblées sur le soutien direct à l'emploi et à l'activité économique auraient dû être reconsidérées.

La prudence, qui était compréhensible dans des circonstances exceptionnelles, s'est malheureusement transformée en une sorte de cavalerie budgétaire d'une année sur l'autre : une partie des crédits non consommés aurait très bien pu être annulée.

En tout état de cause, je tiens à saluer le travail approfondi réalisé par tous les rapporteurs spéciaux de la commission des finances, qui ont analysé très précisément l'exécution de chaque mission budgétaire en cette année particulière et pointé les améliorations qui devront y être apportées.

au contrôle d'Albéric de Montgolfier et de Claude Nougein, qui s'alarment de l'énorme sous-consommation des crédits de la mission « Action et transformation publiques » ; ou encore au rapport que Christian Klinger a consacré à la mission « Santé », montrant la confusion des rôles entre État et sécurité sociale dans la gestion de la lutte contre le covid-19, un an après le transfert de l'agence Santé publique France vers le budget de la sécurité sociale. À l'instar de la Cour des comptes, le Gouvernement plaide pour que le Parlement se penche davantage sur l'évaluation de la loi de finances : je ne doute pas qu'il aura à coeur de tenir compte de ces observations pour le prochain

particulièrement concernées par la transition écologique et durement frappées par la crise, qu'il s'agisse du logement, de l'écologie, des transports terrestres ou aériens, en auditionnant les ministres chargés de ces portefeuilles. Nous espérons que les nombreuses observations que nous avons pu formuler ne resteront pas sans suite.

nous avons appris lundi dernier que la croissance était réévaluée à 6 %, ce que le ministère des finances n'avait semble-t-il pas anticipé dans ses documents budgétaires, la correction ayant été faite aujourd'hui même. Nous savons maintenant, grâce à la dernière allocution du chef de l'État, que s'annoncent un nouveau plan d'investissement, un revenu d'engagement pour les jeunes et d'autres mesures encore

S'il est un domaine où cet effet de loupe a été spectaculaire, c'est bien celui des finances sociales. La construction de notre protection sociale a certes donné une large place aux partenaires sociaux, même si l'État n'était jamais très loin.

D'autre part, la sécurité sociale n'est plus le lieu des seules assurances sociales, elle est le bras armé de l'intervention de l'État dans le domaine social. Monsieur le ministre, face à ce constat, nous avons un désaccord de fond sur ce que doit être l'intervention du Parlement. Si le Parlement s'est un temps effacé au profit de la démocratie sociale, ce ne sont pas les partenaires sociaux qui occupent cet espace, c'est bien le Gouvernement, laissé libre d'agir à sa guise dès lors que la sécurité sociale finance ses interventions. Ainsi, en 2021 pas plus qu'en 2020, nous n'aurons de projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Entre l'effondrement des recettes, l'insuffisance de la provision pour les tests comme pour les vaccins et les nouvelles mesures du Ségur, ce ne sont pourtant pas les motifs qui manquaient.

Face à plus de 30 milliards d'euros de déficit de l'assurance maladie, quelle stratégie privilégier à l'avenir ? Je doute que notre débat d'aujourd'hui permette de répondre à cette question.

prises dans l'urgence pour éteindre l'incendie de l'hôpital, puis du médico-social, ne dessinent pas les contours d'une stratégie claire ni même de priorités, qu'il s'agisse de l'attractivité des métiers, de l'accompagnement des carrières, de l'évolution des statuts ou encore des organisations. Si la crise a révélé les vulnérabilités des services de réanimation, on peinerait ainsi à trouver dans le Ségur les éléments d'un changement structurel. sujet des retraites, les objectifs sont plus clairs. S'ils avaient été formulés en ces termes et non sous la forme d'une grande réforme cérébrale censée ne rien changer pour personne tout en étant plus juste pour tous, nous aurions certainement progressé collectivement.

Là aussi, l'État devra intervenir et nous serions curieux de savoir sous quelle forme. Bien sûr, il est encore trop tôt pour prendre les mesures correctrices nécessaires à une amélioration des comptes sociaux. En revanche, il est grand temps d'y réfléchir et, à tout le moins, de les esquisser. C'est en principe l'objectif assigné au débat d'orientation des finances publiques. Ces dernières ne pourront plus très longtemps être gérées au fil de l'eau,

Mes chers collègues, je vous rappelle que, si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble du projet de loi, dans la mesure où tous les articles qui le composent auraient été rejetés. Or, en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit sur l'ensemble du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020. En conséquence, l'article 8 va être mis aux voix par scrutin public.

des comptes de l'année 2020 ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, le projet de loi n'est pas adopté.

par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

l'amendement n° 709. L'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà un droit de communication des données nécessaires à l'instruction d'une demande de RSA, à sa liquidation et à son contrôle, ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion. La nouvelle rédaction de la commission autorise désormais le président du conseil départemental à demander à tout bénéficiaire du RSA les documents et informations nécessaires pour contrôler la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore ses ressources. Enfin, l'article prévoit que, en cas de refus de communication de ces documents, le président du conseil départemental peut décider de suspendre le versement du RSA.

aux personnes précaires. La précarité a explosé avec la crise sanitaire et vous faites le choix de contrôler encore plus durement les demandes de RSA ! Je rappelle que 36 % des personnes y ayant droit renoncent même à demander cette aide sociale. Par cet

l'amendement n° 1258. Depuis plusieurs années, les dispositifs de contrôle et de sanction se renforcent pour démasquer les fraudeurs parmi les plus précaires.

De même, alors que l'argument avancé est parfois économique, aucune étude n'a été réalisée pour calculer les économies pour les finances publiques que permettraient ces dispositifs de contrôle, au regard de leur coût réel. Nous vivons une crise majeure, qui exige que les organismes sociaux jettent toutes leurs forces dans la lutte contre la pauvreté et pour la réinsertion sociale

En effet, les départements disposent déjà de la compétence du contrôle du service du RSA et de la lutte contre la fraude, au même titre que les organismes de sécurité sociale. La loi leur permet de solliciter toute pièce permettant de vérifier les données des allocataires auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. Les conventions signées entre les départements et les caisses de sécurité sociale permettent de partager l'effort de lutte contre la fraude- car il faut bien lutter contre la fraude ! -, en s'appuyant sur les compétences respectives. Le respect de la vie privée et la préservation des données personnelles imposent que seules les données utiles puissent être partagées. Les pièces personnelles des bénéficiaires sont vérifiées par les caisses de sécurité sociale lors du dépôt de la demande ainsi que lors des contrôles. Cette vérification étant déjà réalisée, permettre aux conseils départementaux de déroger au secret professionnel, principe encadré par la loi, et de disposer de données personnelles non nécessaires à l'insertion sociale et professionnelle

La sollicitation directe auprès des bénéficiaires du RSA de documents justificatifs permettant de vérifier leurs droits à prestation est une prérogative des caisses d'allocations familiales. Pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil départemental dispose, cependant, à l'égard des administrations publiques et des caisses de sécurité sociale, d'un droit de communication des données relatives aux bénéficiaires. auditionné les représentants -considèrent qu'ils ne disposent pas, à l'heure actuelle, de moyens suffisants pour conduire une politique de contrôle efficace. C'est pourquoi, sur l'initiative de Sabine Drexler, la commission des affaires sociales a inséré l'article 35, qui autorise le président du conseil départemental à demander à tout bénéficiaire du RSA les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l'exactitude de ses déclarations. Cet article prévoit également la possibilité, pour le président du conseil départemental, de décider de la suspension du versement du RSA lorsque le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés. À titre personnel, je considère que, en matière d'insertion des bénéficiaires du RSA- ce sont en général des personnes qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé -, le contrôle et les sanctions ne sont pas toujours les instruments les plus efficaces.

est d'être rigoureux dans l'attribution de cette prestation.

Monsieur Savary, monsieur Segouin, vous supposez que l'instruction des demandes de RSA n'est pas rigoureuse, puisque vous défendez l'introduction d'un

d'autant mieux que bon nombre de départements ont renforcé les moyens de ces services. Vous nous dites que vous avez déjà mis en oeuvre des dispositifs de contrôle efficaces, si

et Mme Gatel, au nom de la commission des lois, instaure une possibilité de contrôle des déclarations des bénéficiaires du RSA par le président du conseil départemental. Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet article, notamment en supprimant la mention inappropriée

pleinement leurs responsabilités, et d'améliorer la procédure de sanction actuelle, qui manque de souplesse et qui doit être mieux adaptée à la nature du non-respect des obligations du bénéficiaire. Le RSA est bien un revenu de solidarité active : ce n'est pas une rente. Le but est bien de rencontrer les personnes bénéficiaires pour les guider et les aider à se réinsérer par le travail.

eux, seuls 6 % des logements en France sont adaptés à la vie quotidienne des personnes en perte d'autonomie. L'habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale, dit API, aussi appelé «

Dans un rapport rendu au mois de juin 2020, MM. Denis Piveteau et Jacques Wolfrom notaient le rôle central que devra nécessairement jouer, à l'échelon local, la collectivité territoriale départementale. Ils précisaient également que ces logements accompagnés, partagés et insérés dans la vie locale n'avaient de sens que s'ils s'inscrivaient dans une démarche d'habitat et d'urbanisme très générale. C'est pourquoi je me réjouis que ce projet de loi prévoie en son article 36 la faculté pour le département de coordonner le développement de l'habitat inclusif et l'adaptation du logement au vieillissement de la population,

aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé et assorti d'un projet de vie sociale défini par un cahier des charges national.

l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Alain Milon, cette compétence a été assortie de leviers plus opérationnels. Cela va dans le bon sens et c'est cohérent avec l'aide à la vie partagée que les règlements départementaux d'aide sociale

est formellement alloué par la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, afin d'éviter que les appels à projets lancés par les ARS puissent avoir lieu sans que les départements soient mis dans la boucle.

aux personnes versées par les départements, désormais responsables de la coordination des acteurs. Sous réserve que le Gouvernement confirme la faisabilité du dispositif, la commission émet un avis favorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement

Plus précisément, il s'agit de donner une base légale à l'organisation de l'exercice des missions relevant des maisons territoriales de l'autonomie. En effet, si Saint-Barthélemy peut créer une maison territoriale de l'autonomie au titre de la compétence départementale, le droit commun n'est pas adapté à la taille de la collectivité. Il ne tient pas compte de l'absence de certains collèges composant les organes participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques d'autonomie, tels que le conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie

En effet, pour la prise en charge de la politique en faveur de l'autonomie des personnes handicapées et âgées, la création d'un groupement d'intérêt public est démesurée au regard de la taille du territoire. Actuellement, l'instruction des demandes d'aide au profit des personnes handicapées est menée par l'équipe pluridisciplinaire du conseil départemental de la Guadeloupe, en lien avec le service de la collectivité en charge de la cohésion sociale. Celui-ci assure, par ailleurs, l'ensemble des missions relatives à l'autonomie des personnes âgées. Il s'agit donc de permettre à Saint-Barthélemy de mettre pleinement en oeuvre la politique d'autonomie des personnes handicapées, en permettant que la maison territoriale de l'autonomie déroge au statut de groupement d'intérêt public au profit d'un service de la collectivité.

dans le code de l'action sociale et des familles la morphologie du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, pour l'adapter à la situation particulière de Saint-Barthélemy. En effet, la collectivité ne dispose pas de représentants pour tous les services actuellement prévus dans le code de l'action sociale et des familles pour composer ce conseil dans les départements métropolitains. à prévoir la base légale nécessaire à la création d'une maison territoriale de l'autonomie, équivalent des maisons départementales de l'autonomie qui regroupent les services départementaux destinés aux personnes âgées et la maison départementale

Sans doute faudrait-il, en outre, que la situation de Saint-Martin soit également prise en compte. La commission a donc souhaité avoir l'avis du Gouvernement sur la robustesse technique de l'amendement.

la forme d'un groupement d'intérêt public une maison départementale des personnes handicapées. Par ailleurs, une réflexion est actuellement engagée avec la collectivité de Saint-Martin, dont les problématiques, qu'il s'agisse de l'éloignement ou de l'insularité, sont communes

Il nous a donc paru pertinent de chercher des solutions pour faciliter la venue des étudiants au sein de ces territoires. L'amendement qui tendait à instaurer une telle expérimentation a été malheureusement jugé irrecevable. Les mesures visant à faciliter la location de logements à des publics cibles sont essentielles pour assurer le dynamisme des territoires et l'inclusion de tous en leur sein. Tel est l'objet de cet article et tel était aussi l'objet de notre amendement, monsieur le rapporteur

et la dépendance s'y installe de façon plus précoce que dans le territoire hexagonal. La perte d'autonomie se cumule avec un taux de pauvreté de la population âgée qui est trois fois supérieur à celui de l'Hexagone.

rendre applicables certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux foyers logement dans certains territoires ultramarins. Il existe une grande convergence de vues en faveur du développement des résidences autonomie dans les outre-mer, où le vieillissement de la population sera globalement important et assez rapide. les échanges que j'ai eus avec le ministère des solidarités et de la santé indiquent qu'une telle disposition ne suffirait pas, sans que les autres modifications opérées aient été exposées clairement. En toute hypothèse,

communautés urbaines ne puissent pas exercer une compétence d'action sociale ni créer un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Actuellement, seules les communautés de communes et et d'agglomération en ont la possibilité. Nous estimons que l'extension proposée rendrait illisibles les spécificités de certaines communes sans leur laisser la possibilité démocratique de se faire entendre. Elle renforcerait en outre les inégalités intra-départementales. Plus globalement, nous sommes défavorables au transfert de l'action sociale des communes aux regroupements de communes, car cela éloignerait les administrés des centres d'action sociale. Or, dans ce secteur, nous connaissons les difficultés de mobilité des publics précaires pour se

à conserver le pilotage de l'action sociale dans les collectivités. Quel

de se doter d'un centre intercommunal d'action sociale. Actuellement, les communautés de communes et d'agglomération sont les seules qui disposent de cette compétence, de façon obligatoire ou optionnelle. Elles bénéficient à ce titre de la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, qui est indispensable pour créer un CIAS. Il convient de reconnaître aux communautés urbaines et aux métropoles la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, afin de répondre au mieux à de nouvelles problématiques sociales complexes et polymorphes. Il s'agit de rendre compatible l'exigence de proximité avec des politiques sociales ambitieuses. L'objectif est de doter les territoires de plusieurs leviers de développement en conformité avec la logique de mutualisation.

Merci ? Cet amendement a pour objet d'attribuer aux communautés urbaines et aux métropoles la compétence obligatoire d'action sociale d'intérêt communautaire et de fonder ainsi la possibilité de créer un centre

celles qui exercent une compétence d'action sociale de manière facultative auraient la possibilité de créer un CIAS. Toutefois, il pourrait être envisagé de confier une compétence obligatoire d'action sociale d'intérêt communautaire aux métropoles et communautés urbaines, afin de leur permettre de remplir les conditions prévues à l'article L.

des suffrages exprimés par celle de l'unanimité pour les décisions concernant la création d'un centre intercommunal d'action sociale, au sein d'une métropole ou d'une communauté urbaine.

aux départements, en cohérence avec les missions des départements, responsables du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et de la mise en oeuvre des mesures administratives et judiciaires de protection de l'enfance. Les règles applicables au statut de pupille de l'État ne seront pas modifiées. En plus de la gestion du parcours des pupilles qu'il assume déjà aujourd'hui- je tiens à le préciser -, le département se verra confier leur tutelle. La mesure permet ainsi de renforcer le suivi de proximité des pupilles, en confiant au département la fonction de tuteur. exercera ainsi au plus près des besoins de l'enfant les actes usuels de l'autorité parentale aux côtés du conseil de famille. Afin de garantir un équilibre en faveur des droits des mineurs admis comme pupilles de l'État, sous la responsabilité du département, il est proposé que les représentants du département ne soient plus membres du conseil de famille. En outre, avant toute décision du président du conseil départemental relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'État, l'accord du conseil de famille devra être recueilli. Le rôle de l'État est donc garanti et le rôle du département sur des compétences qu'il exerce déjà est conforté.

sa place dans le projet de loi relatif à la protection des enfants, que nous examinerons prochainement et qui a déjà été discuté à l'Assemblée nationale. Elle a, en outre, considéré que les conditions d'application de ce transfert dans l'ensemble des départements, notamment pour ce qui est des moyens, n'étaient pas suffisamment précisées. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement tendant

que les enfants ne soient pas sous la responsabilité pleine et entière du département. Même si celui-ci a la responsabilité du parcours de l'enfant,

dans le placement d'enfants qui sont délaissés. Or le délaissement parental est aussi un sujet important pour les départements. Enfin, je veux insister sur le fait que cet article ne garantit nullement que les pupilles bénéficieront d'un traitement égal sur tous les territoires. Il suffit de se référer au dernier rapport de

En commission des affaires sociales, M. le rapporteur pour avis a très justement rappelé que la France avait conclu, ces dernières années, de tels accords avec l'ensemble des pays limitrophes de l'Hexagone, à l'exception de l'Italie. Il a également rappelé, ce dont je lui sais gré, qu'il n'existait pas à ce jour d'accord avec un pays voisin d'un territoire d'outre-mer. d'outre-mer. Si la signature d'un accord-cadre de coopération sanitaire ne conditionne pas, sur le terrain, l'existence de formes de coopération, les exemples allemands, belges, ou espagnols sont là pour nous montrer tout l'intérêt que peut avoir ce type d'entente. Il est évident que de tels accords trouveraient parfaitement leur place dans la Caraïbe, en particulier aux Antilles, dont vous connaissez la géographie autant que le potentiel en matière de santé, C'est pourquoi il me semble, même si ce n'est pas tout à fait l'objet de cet article, que le Gouvernement et le Sénat gagneraient à approfondir ce sujet. Par ailleurs, madame la ministre, le Gouvernement a peut-être des éléments à nous communiquer à ce sujet dès aujourd'hui.

Cet amendement vise à faciliter la prise en charge des problématiques de santé à une échelle transfrontalière, en offrant la possibilité d'élaborer des contrats locaux de santé transfrontaliers.

ne nous semble pas pertinent de prévoir la nécessité de tels contrats locaux de santé ni, surtout, de lever la condition d'existence d'un accord international. La santé relève bien d'une compétence de l'État : c'est à celui-ci qu'il revient d'organiser avec le pays limitrophe les conditions et les modalités de la coopération y associer les collectivités étrangères, ce qui peut sembler pertinent, laisse cependant entendre que les collectivités sont toutes compétentes en matière de santé, en France comme à l'étranger, ce qui n'est pas sûr. Par conséquent, la commission demande le retrait

De plus, l'enregistrement des données personnelles des enfants à d'autres fins que celles qui sont liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations unies. À l'inverse d'une généralisation du recours à ces fichiers, nous considérons qu'il est absolument nécessaire de supprimer la possibilité pour les conseils départementaux de recourir au fichier national biométrique d'appui à l'évaluation de la minorité.

écartée lorsque celle-ci n'est pas manifeste. Il s'agit d'un principe absolu ! De plus, comme l'indique le Conseil national des barreaux, la création de ce fichier est critiquable, dès lors qu'il suppose pour sa mise en oeuvre le lancement d'investigations dont la durée d'accomplissement est incompatible

alors que le projet de loi relatif à la protection des enfants a été soumis au Parlement le 16 juin dernier et qu'un rapport de contrôle sur les mineurs non accompagnés est en cours d'élaboration au Sénat, nous nous étonnons de la précipitation du Gouvernement à vouloir légiférer en la matière, particulièrement au sein au sein d'un projet de loi relatif à l'organisation territoriale de notre République. Il convient donc, selon nous, de supprimer sans plus attendre cet article.

devant un juge des enfants. Faute de renforcer les budgets alloués aux départements, une telle proposition, inefficace et démagogique, n'apporte aucune protection pour les enfants et les jeunes majeurs. En imposant l'utilisation de ce fichier, le Gouvernement veut tordre le bras aux derniers départements qui refusent de confondre protection de l'enfance et lutte contre l'immigration, en les pénalisant financièrement. Cet article fait passer la question migratoire avant les droits de l'enfant et met à mal la règle de présomption de minorité, en passant d'une évaluation en cas de doute à une évaluation sauf en cas de minorité manifeste. Pour ces raisons, le groupe SER propose également la suppression de cet article.

le nomadisme de certaines personnes qui ne sont pas forcément mineures, mais vont demander à être reconnues comme telles dans plusieurs départements, alors même que leur

? Comme chacun le sait, c'est le Gouvernement qui a proposé la mise en place du fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, le fameux fichier AEM, qui a pour objectif de permettre à un département recevant une demande de reconnaissance de minorité d'avoir connaissance des décisions déjà prises par d'autres départements à l'égard du même demandeur. Il s'agit simplement de canaliser le phénomène des demandes multiples, chaque département demeurant responsable de ses décisions. Je rappelle également que la procédure de présentation en préfecture aux fins d'enregistrement du demandeur dans le fichier ne porte que sur les demandeurs dont la minorité n'est pas manifeste.

Face à de tels sujets, on ne peut pas s'en sortir en disant simplement que c'est un sujet sensible. Cela concerne des enfants.

pourraient consacrer leur énergie à mettre en oeuvre des solutions plutôt qu'à répéter des procédures faites ailleurs. Rappelons aussi que le recours à ce fichier ne vaut pas déclaration de minorité ou de majorité.

car il s'agit bien là de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, seuls 30 % des jeunes qui demandent la reconnaissance de leur minorité la voient reconnue lors de l'évaluation par les départements

services départementaux d'aide sociale à l'enfance et qui formulent un recours auprès du juge pour enfant voient leur minorité reconnue par l'autorité judiciaire.

international, lequel consacre le principe de présomption de minorité de manière claire, tant dans la jurisprudence que dans les textes internationaux. en 2019, trois décisions du Comité des droits de l'enfant des Nations unies rappellent que, jusqu'à la décision judiciaire définitive, la personne doit être protégée et traitée comme un enfant.

par le Comité des droits de l'enfant des Nations unies. Nous avons déposé un amendement en ce sens, qui a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution- c'est une preuve de la non-application du principe de présomption de minorité. Nous le regrettons comme une occasion manquée pour la France de se conformer sans ambiguïté à la Convention internationale

L'article 39 prévoit notamment que le conseil départemental puisse demander à l'autorité judiciaire de recourir aux tests osseux dans le cadre de l'évaluation de minorité. de minorité. Or les méthodes d'évaluation de la minorité doivent découler en priorité de l'entretien pluridisciplinaire et non de la comparaison d'éléments fondés sur la seule apparence et sur les tests osseux, qui sont contestables quant à leur fiabilité scientifique et intolérables d'un point de vue éthique. Par conséquent, il est impératif de recourir à d'autres méthodes

En cas de persistance d'un doute dans la détermination de la minorité, celui-ci doit profiter aux jeunes. Tout examen médico-légal doit être interdit : la santé qui soigne n'a pas vocation à être un outil à expulsion. Il est donc urgent de mettre fin aux tests osseux, plus globalement aux ingérences du ministère de l'intérieur dans le dispositif d'évaluation médicale, ainsi que de restaurer la tutelle du ministère de la santé. De plus, il est nécessaire que l'évaluation de minorité soit réalisée par une équipe pluridisciplinaire afin d'écarter toute coopération entre le conseil départemental et le préfet. C'est pourquoi

dans sa décision du 21 mars 2019. Je rappelle que ces tests osseux ne sont décidés que par l'autorité judiciaire, après accord de l'intéressé. On sait également que les résultats d'examen font mention de la marge d'erreur et ne peuvent permettre à eux seuls de déterminer que la personne est mineure. Le reste du dispositif, notamment les entretiens conduits par le conseil départemental, est maintenu et reste absolument nécessaire. La commission émet donc un avis défavorable

Mme Raymonde Poncet Monge. L'article 47 du code civil dispose que les documents d'état civil, même étrangers, font foi pour établir l'identité d'un individu devant les autorités françaises. De même, l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant consacre le droit à l'identité du mineur en prévoyant la reconnaissance des documents d'état civil présentés. De même, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies affirme que les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire. Ainsi, les documents d'état civil étrangers doivent être présumés valides et cette présomption est juridiquement établie. Pourtant, bien souvent, les mineurs non accompagnés sont soumis à d'autres méthodes d'évaluation de leur minorité, alors même qu'ils ont présenté un document d'état civil qui n'a pas été contesté. contesté. On a parlé des tests osseux, considérés comme faisant foi, alors même que ce test possède un grand degré d'incertitude. Cela conduit, aujourd'hui, à des vices de procédure sur lesquels les cours administratives d'appel multiplient les jurisprudences. Deux circulaires encadrent pourtant les pratiques. La circulaire du 1 avril 2003

en précisant le rôle du département et en posant des conditions à la saisine du préfet chargé de mettre en oeuvre les vérifications nécessaires à l'authenticité des documents. Pourtant, alors même que ces textes précisent que ces saisines ne peuvent jamais revêtir un caractère systématique, force est de constater que les pratiques restent parfois entachées d'irrégularités. Cet amendement de clarification vise à faire entrer dans la loi les dispositions de la circulaire de 2016 précitée, qui précise le rôle des départements dans les procédures de vérification.

l'avis de la commission ? Il faut distinguer l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il n'est pas question ici de remettre en cause, et des procédures qui découlent de dispositions législatives, dans cette situation comme dans d'autres. chère collègue, il est difficile de porter une appréciation véritablement juridique sur la notion de documents non formellement contestés.

à la vérification ou à l'authentification des documents d'état civil est déjà prévue à l'alinéa 8 de l'article 39 et est déjà facultative. Ce point-là est donc largement satisfait. satisfait. En outre, demander au conseil départemental de vérifier la reconstitution d'un état civil ne relève pas de son champ de compétences. Il me semble que le département doit se concentrer sur les solutions à mettre en oeuvre

dans un pays éloigné demande un délai souvent assez long, de l'ordre de plusieurs mois, qui n'est pas compatible avec les délais très brefs qui s'imposent au processus d'évaluation de la minorité. En effet, ce processus doit normalement être mené à son terme durant la période de mise à l'abri de la personne se disant mineur non accompagné, c'est-à-dire cinq jours. Ce n'est pas très compatible avec la recherche de papiers. C'est pourquoi ces démarches ne peuvent être utilement entreprises que durant la période de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance. En d'autres termes, le jeune est là et il s'agit de savoir s'il est mineur et doit

cela, le président du conseil départemental décidait du recours ou non à ce fichier par ses services, en sollicitant ou non le concours du préfet.

Il n'existe pas de statut juridique propre aux mineurs isolés étrangers. Ces derniers se trouvent donc au croisement de celui qui relève du droit des étrangers, celui qui relève de l'enfance en danger et du dispositif français de protection de l'enfance, qui ne pose aucune condition de nationalité. C'est le statut d'enfant qui devrait prévaloir pour ces personnes et non le statut d'étranger, conformément aux engagements de la France au titre de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est ce que le groupe Demander une protection n'est pas simple. Cette démarche se révèle d'autant plus difficile lorsque les départements choisissent de mettre en place un processus où l'enfant devra d'abord aller au commissariat

Cette logique répressive et de défiance grandissante à l'égard de ces enfants en grande précarité et vulnérabilité devrait définitivement être renversée et cesser. Quel

au mois de juillet 2019, dans une autre QPC, que son usage n'était pas contraire à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur

Tout cela est bien joli, mais il faudra tout de même revenir, un jour ou l'autre, au principe fondamental de ce qui fait la nationalité. La Cimade, cette organisation militante, affirme que l'enregistrement des données personnelles des enfants à d'autres fins que celles qui sont liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du Comité des droits de l'enfant unies. Si je comprends bien, dans le « nouveau monde » de ce Gouvernement, on pourrait ficher un enfant mineur parce qu'il n'est pas vacciné et, à cet autoritarisme, les communistes ajouteraient le laxisme migratoire. Pour eux, on ne pourrait pas ficher des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des clandestins, dans le cadre d'une politique de contrôle des flux migratoires. Il me semble urgent de revoir les priorités et les réalités. En France, les Français de tous âges vivent libres et protégés, particulièrement les mineurs. C'était tout du moins le cas jusqu'à lundi,

l'un de ces mots qui rassemblent celles et ceux qui ont combattu ensemble pour la liberté dans notre pays. Vous n'êtes pas les seuls ! C'est l'un de ces mots qui rassemblent celles et ceux qui ont combattu l'occupation dans notre pays pour rétablir la République au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce mot qui rassemble celles et ceux qui, aujourd'hui, se battent pour le bien-vivre, pour la fraternité, pour le progrès social. Vous pouvez

de contredire la décision d'un conseil départemental sur la minorité d'une personne se présentant comme MNA. Cela porte atteinte au principe constitutionnel d'indépendance de la justice.

amendement. La décision de retenir l'état de minorité relève de la seule appréciation du juge, qui se fonde sur un faisceau d'indices constitué des déclarations du jeune en audience, de l'évaluation réalisée par les services du conseil départemental, des documents d'identité présentés et, le cas échéant, des conclusions d'un examen radiologique que seule l'autorité judiciaire peut ordonner. L'évaluation effectuée par le conseil départemental est un élément essentiel de sa prise de décision, mais ne peut se substituer à la décision juridictionnelle.

à la fonction publique territoriale et non plus à la fonction publique hospitalière, comme c'est le cas aujourd'hui. Si nous pouvons partager la volonté de revenir sur l'éclatement des compétences entre les ministères et les collectivités, afin de renforcer les services de la protection de l'enfance, ce transfert inquiète légitimement les directrices et directeurs de l'enfance et de la famille.

pour leur rattachement à la politique familiale du ministère, qui doit primer sur les aspects départementaux. Le rattachement des directeurs des établissements de la protection de l'enfance à un corps national commun au directeur des secteurs social, sanitaire et médico-social constitue un élément fort d'expertise, de partage et d'harmonisation des pratiques professionnelles sur l'ensemble du territoire national. Je rappelle, à ce titre, que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ont rendu un avis défavorable Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 40 et l'ouverture de véritables négociations avec les directrices et directeurs de l'enfance et de la famille pour améliorer la coordination des structures en faveur de l'action sociale, qui est

sur cet amendement. Nous nous fixons tous ici, le Gouvernement comme chacun d'entre nous sur ces travées, un objectif d'efficacité : rendre le meilleur service, jusqu'au dernier kilomètre, sur l'ensemble des compétences. Il existe des compétences partagées entre l'État et les collectivités ; c'est le cas de la santé. Je rappelle que les lois de décentralisation ont confié aux départements la protection de l'enfance et que les départements exercent cette compétence d'une manière extrêmement satisfaisante. Aussi, chacun d'entre nous ne peut que leur rendre hommage, comme nous devons rendre hommage aux personnels qui travaillent dans ces établissements autour de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, mes chers collègues, permettez-moi d'être factuelle et de présenter la situation. Aujourd'hui, le le président du conseil départemental et son département ont la responsabilité de la protection de l'enfant. C'est donc le département qui est comptable du service rendu, de son efficacité et du fait qu'il trouve des solutions pour l'ensemble des enfants.

comment ne pas accepter le rattachement de ces personnels aux départements ? Nous avons eu l'exemple de transferts de personnel d'État vers les collectivités, qui se sont plutôt bien passés. Je rappelle, en rendant hommage à ces personnels,

supérieurs à ceux qu'ils pourraient avoir dans la fonction publique territoriale. En outre, chacun sait que les avancements dans la fonction territoriale sont plus aisés et que la difficulté que rencontre un département

en matière d'action sociale, en dépit du rôle de chef de file que la loi confère au département et au détriment de l'efficacité des politiques menées et de leur lisibilité pour les usagers.

La principale, qui fait l'objet d'un large consensus parmi les départements, est la création d'une agence départementale des solidarités, placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l'ensemble des acteurs. La parole est à M.

rendu public le 2 juillet. La mission d'inspection y préconise de donner au conseil départemental une compétence supplémentaire en matière de repérage des violences conjugales, y compris en l'absence de maltraitance infantile. Considérant qu'il n'y a pas de temps à perdre,

Mme la ministre.

de protection de l'enfance. Toutefois, si les conseils départementaux ont un rôle à jouer dans le repérage des violences au sein des couples, leur mission première doit demeurer la protection de l'enfant. Leur action doit être centrée sur les besoins fondamentaux de l'enfant et sur la capacité de ses parents je vous remercie

qui traduit les cinquante propositions du Sénat présentées le 2 juillet 2020 à la suite des travaux de la commission des lois et de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur l'avenir de la décentralisation. Cet amendement vise à conforter le pouvoir des départements en matière de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les directeurs seraient désormais nommés par le président du conseil départemental. Après près de quarante ans de décentralisation, l'adoption de cet amendement permettrait de donner à la libre administration des collectivités territoriales sa pleine mesure, pour une plus grande efficacité de l'action publique. La parole est à M.

sur les amendements n 578 et 580, le Gouvernement est défavorable à un tel ajout.

la pandémie, il y a eu des collectivités, quelles qu'elles soient- des départements, des régions et des villes -, pour venir en aide aux étudiants, qui se trouvaient dans des situations parfois

mission à laquelle est censée participer l'ensemble de la communauté éducative. La Cour des comptes, dans un rapport de 2020, a encore étrillé la santé scolaire, mais elle estime que ses dysfonctionnements tiendraient moins à un manque de moyens et de personnel qu'aux « failles de son organisation et à son défaut de pilotage Cette situation s'explique « par l'opacité de l'exercice des activités et le cloisonnement des personnels », qui ont beaucoup de mal à travailler ensemble et refusent tout lien hiérarchique entre eux. une performance très en deçà des objectifs de dépistages obligatoires, due à une organisation défaillante ». Entre 2013 et 2018, le taux de réalisation de la visite de la sixième année de l'enfant par les médecins scolaires, en principe généralisée et déterminante au début des apprentissages scolaires, aurait chuté de 26 %, taux déjà très bas, à 18 % ! L'éducation nationale a vraisemblablement failli à sa mission légale de promotion de la santé scolaire. Aussi souhaitons-nous confier cette mission aux départements. Ceux-ci ont déjà une compétence obligatoire en matière de protection sanitaire et sociale des enfants. Il y aurait ainsi une logique à confier ces deux missions complémentaires à cette même autorité. À défaut d'un transfert légal, nous souhaitons que le Gouvernement rende un rapport au Parlement sur le sujet. Quel est l'avis de la commission

dans les décisions d'ouvrir ou de fermer des écoles ou des classes, tout particulièrement en milieu rural. Aujourd'hui, la loi

pour fermer des classes ou regrouper des écoles. Et, madame la rapporteure, ne soyez pas du tout inquiète quant à mes capacités de mobiliser les maires de mon département pour s'opposer aux fermetures de classes. Je le fais plus souvent qu'à mon tour

La séance est suspendue.